pas parmi les établissements d'enseignement qui sont expressément exonérés de la taxe sur les bureaux en Île-de-France. Pourtant, leur activité d'enseignement présente un caractère d'intérêt général indéniable et les conditions d'exercice de cette activité sont directement comparables à celles des établissements d'enseignement qui sont, eux, exonérés.

Un de ses points clés est notamment le développement de ces centres de formation pour apprentis, afin de pouvoir répondre aux besoins en compétences des entreprises. Dans ces conditions, il va sans dire que cet impôt va à l'encontre des objectifs affichés en la matière par le Gouvernement. L'apprentissage concourt aux objectifs généraux de la Nation, il est donc légitime que les locaux des CFA ne soient pas assimilables à des locaux commerciaux. Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette inégalité de traitement, en exonérant les CFA de la taxe sur les bureaux applicable en Île-de-France.

pondéreux. Or l'un des freins à l'émergence du fret ferroviaire comme une solution pérenne pour acheminer les marchandises en zone urbaine réside dans la difficulté à trouver un équilibre économique pour l'investissement dans les terminaux ferroviaires urbains, qui constituent le point d'arrivée des marchandises avant la livraison du ou des derniers kilomètres. Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, les auteurs de cet amendement proposent d'exonérer

compétent de collectivité locale. La répartition de cette redevance est aujourd'hui calculée au seul prorata des enjeux réalisés sur les courses hippiques organisées par chaque hippodrome. Cette méthode de calcul privilégie certains hippodromes, sur lesquels se courent des courses premium supports de Quinté plus et n'est pas corrélée au nombre de réunions de courses organisées réellement par ces hippodromes. En pratique, 80 % de l'enveloppe sont redistribués à 25 EPCI sur les 193 qui possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels et seuls 4 EPCI atteignent le plafond de 772 000 euros. 45 % des EPCI concernés touchent une redevance inférieure à 1 000 euros. Celle-ci, de par son montant, n'est pas toujours identifiée, et en tout cas pas identifiée comme un retour issu de l'activité de l'hippodrome. Or nous le savons, en tant qu'élus de territoires, ces hippodromes jouent un rôle majeur en matière d'animation du territoire. Il importe donc que l'ensemble de ces enjeux y participe d'une manière plus équitable et soit réparti sur le territoire. C'est pourquoi affecter 25 % de l'enveloppe au prorata du nombre de réunions de courses organisées et baisser le seuil maximal par collectivité permettraient cette répartition et respecteraient mieux l'implication des collectivités. Sur un total de 193 collectivités, cette méthode entraînerait une augmentation de la redevance dans 173 cas. Le deuxième volet de cet amendement aborde la question de la compétence. Depuis la compétence. Depuis 2010, cette redevance a été affectée tour à tour aux communes puis aux EPCI. Plutôt que d'imposer une affectation fixe à l'un ou à l'autre de ces niveaux avec de fréquentes complications de réaffectation, il serait préférable d'allouer cette redevance au niveau qui est effectivement attributaire de la compétence. Je rappelle que la compétence « hippodromes » n'est pas obligatoire. Elle est donc communale, à moins d'un transfert à l'EPCI.

Loisier, vise à rétablir une certaine équité au profit des territoires ruraux. On constate que ce prélèvement sur les enjeux hippiques, dans la limite de 772 000 euros par EPCI, est essentiellement réparti sur 12 % des territoires qui en concentrent 80 % des montants, ce qui est assez inéquitable. En effet, celui-ci est calculé en fonction des

par un EPCI siège d'un ou de plusieurs hippodromes et d'introduire un nouveau critère de répartition, à savoir 75 % dans la limite des enjeux et 25 % en fonction du nombre de réunions de courses organisées par les hippodromes.

Effectivement, 4 collectivités sur 193 connaîtront une diminution, tandis que la grande majorité bénéficiera d'une hausse

bénéfices alors qu'ils n'ont pas spécifiquement une compétence en matière de gestion de ces équipements.

pour certains territoires, au détriment des autres. En effet, le droit existant plafonne le reversement du prélèvement sur les paris hippiques à 772 000 euros par EPCI. L'article prévoit de répartir ce produit à 50 % pour la commune et 50 % pour l'EPCI et divise par deux le plafonnement qui s'appliquerait aux communes et

nous concentrions les moyens sur quelques

marchandises ... Or l'organisation des courses hippiques ne peut être assimilée dans sa globalité à un usage commercial. Seuls quelques espaces isolés peuvent être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales, mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces, qui sont pour leur majeure partie des surfaces naturelles non bâties, notamment les pistes. Plusieurs DDFiP se sont rangées à ces arguments et ont accepté de revoir à la baisse les taxes foncières, comme en attestent les décisions récentes en faveur des hippodromes de Vittel et des Andelys. Les services fiscaux ne peuvent faire valoir des règles différentes selon la seule appréciation des responsables départementaux.

Vous proposez d'imposer à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFPNB, tous les terrains affectés à l'usage des courses hippiques, comme c'est actuellement le cas pour les golfs. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette proposition. Tout d'abord, les terrains hippiques peuvent déjà être soumis à la TFPNB. En effet, seuls les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour les hippodromes, les terrains affectés aux pistes d'entraînement ou de compétition sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties uniquement lorsqu'ils présentent un usage commercial. Dans le cas contraire, ils sont imposables selon le régime du foncier non bâti. Ensuite, le transfert systématique des terrains hippiques exploités commercialement de la TFPB à la TFPNB aurait des conséquences non négligeables. Les valeurs locatives sont plus faibles en foncier non bâti qu'en foncier bâti. Les collectivités percevraient donc une recette foncière plus faible qu'aujourd'hui. Les départements qui ne perçoivent plus de TFPNB ne tireraient alors plus aucune recette des terrains hippiques. Les communes et EPCI subiraient également une perte de cotisation foncière des entreprises,

à imposer le bâtiment donné à bail emphytéotique hospitalier dès lors qu'il serait productif de revenus pour l'emphytéote. En outre, l'exonération ne serait applicable que pendant la durée du bail emphytéotique. À l'issue du bail, le bien redeviendrait la propriété du groupement de coopération sanitaire et serait alors soumis à la taxe foncière. L'amendement de précision de précision n° II-993 participe du même objectif. Peut-être gagnerait-il encore à être amélioré lors de la navette, mais, parmi les deux voies proposées pour atteindre le même objectif, nous souhaitons que la voie choisie par le Gouvernement soit privilégiée.

trois amendements visent à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui seraient confrontés à une baisse imprévisible et exceptionnelle de l'assiette d'une imposition directe locale de prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année en matière de cotisation foncière des entreprises,

En l'état actuel du droit, les opérateurs ayant investi plus tardivement dans la fibre optique ne supporteraient pas les mêmes charges que ceux qui ont été précurseurs dans le déploiement de cette technologie, ce qui créerait une distorsion de concurrence. Pour remédier à cette situation, sans remettre en cause le principe de l'élargissement de l'assiette de l'IFER, cet amendement prévoit, d'une part, de revenir à la tarification prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2017 et, d'autre part, de reporter l'entrée en vigueur de l'imposition à 2022, horizon fixé par le Gouvernement pour atteindre le très haut débit pour tous. Cet amendement serait ainsi en cohérence avec le calendrier de la réforme de la fiscalité locale, un projet de loi

huit années les réseaux FTTH- -de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ou IFER, prévue à l'article 1599 B du code général des impôts,

d'au moins sept ans avec celui de la zone d'investissement privé. Avec un tel système, l'accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut débit ne seront pas pénalisées. Quel est l'avis de la commission ? Ces amendements

l'une des conclusions du groupe de travail sur l'éolien terrestre mis en place par Sébastien Lecornu lorsqu'il était secrétaire d'État, et sur laquelle un consensus avait été trouvé. Deuxièmement, il s'agit simplement de garantir que les communes accueillant des éoliennes pourront percevoir 20 % de l'IFER, quel que soit le régime juridique de leur EPCI, et seulement si elles le souhaitent. Troisièmement, cette disposition ne s'appliquera que pour les projets mis en service après le 1 janvier 2019, afin de ne pas remettre en cause les accords déjà conclus entre les EPCI et les communes d'accueil. Enfin, à ceux qui objecteraient que l'on voudrait créer un cas particulier pour l'IFER éolien par rapport à l'IFER nucléaire, solaire ou autre, j'indique que ce traitement particulier est parfaitement justifié. En effet, parmi les énergies renouvelables, l'éolien terrestre crée des nuisances plus fortes pour la commune d'implantation que les panneaux solaires, par exemple. Personne ne peut le contester. Quant au nucléaire, chacun conviendra que le sujet dépasse très largement celui de l'IFER et qu'il est, du reste, très peu probable que la question de l'implantation de nouvelles centrales dans les territoires qui n'en accueillent pas déjà se pose dans les prochaines années.

l'avis du Gouvernement ? Le Gouvernement est attaché à cet article pour trois raisons. D'abord, les communes sur lesquelles sont implantées les installations éoliennes subissent directement leurs externalités négatives, notamment les nuisances visuelles. Ensuite, l'article 56 préserve un certain équilibre dans la répartition des ressources fiscales entre les communes et les EPCI. En effet, même si les communes membres d'EPCI à fiscalité professionnelle unique et à fiscalité économique unique perçoivent désormais 20 % du produit de l'IFER, elles auront la possibilité de délibérer afin de transférer tout ou partie de cette somme au bénéfice de leur EPCI, afin de lui donner les moyens d'agir. Enfin, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux installations éoliennes construites à compter du 1 janvier 2019 et ne remettent donc pas en cause la répartition du produit des IFER

des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l'horizon de 2030. Dans ce contexte, différents projets sont menés dans les territoires afin de permettre une accélération de leur rythme de développement, tout en garantissant la protection de l'environnement et du cadre de vie. Pour les communes susceptibles d'héberger des parcs éolien ou photovoltaïque, la fiscalité est un enjeu majeur, car elle peut représenter un attrait financier non négligeable. Si l'on peut se réjouir des avancées significatives sur la fiscalité éolienne introduites par un amendement adopté à l'Assemblée nationale, qui permet aux communes accueillant des éoliennes de percevoir jusqu'à 20 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, on peut regretter l'absence de similitude avec le photovoltaïque. Par conséquent, cet amendement vise, d'une part, à corriger cette injustice et, d'autre part, à faire en sorte que cette mesure ne s'applique qu'à partir du 1 janvier 2019, afin de ne pas revenir sur les accords déjà conclus

sur le tarif de la taxe d'aéroport applicable aux passagers en correspondance de 40 % à 65 %, afin de nous donner la possibilité de renforcer la compétitivité des plateformes françaises de correspondance, notamment celles de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Lyon-Saint-Exupéry.

doit permettre à l'État de réaliser une économie de 800 millions d'euros, soit 40 % du montant du crédit d'impôt, et cela au détriment de la réalisation urgente des objectifs de rénovation thermique de l'habitat.

la période, durant laquelle les contribuables domiciliés en France pourront bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. Cela concerne notamment l'acquisition de chaudières à haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques et enfin l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage. Le crédit d'impôt va de 15 % à 30 % de la dépense suivant les types de matériaux.

par le biais d'un crédit d'impôt- c'est ce que l'on appelle la transition énergétique positive. Ce soutien public est d'autant plus légitime que le changement de fenêtres est souvent le point d'entrée dans un parcours de rénovation thermique du logement- on commence par les fenêtres, puis on fait la toiture ou l'isolation extérieure, où les sommes à mobiliser sont naturellement bien plus importantes. Il s'inscrit aussi dans le contexte que chacun connaît de prix élevés de l'énergie. Cet amendement, qui constitue une réponse très concrète aux difficultés que rencontrent les Français pour se chauffer,

Dans le souci d'optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise donc d'intégrer dans le CITE les systèmes de ventilation mécanique contrôlée au taux de 15 %.

et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l'activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique. On rappellera que ce sont les particuliers qui doivent payer la transformation énergétique du secteur de l'habitat, en rénovant leur propre logement. Comment pourront-ils le faire massivement, et plus qu'aujourd'hui, si dans le même temps le Gouvernement n'a de cesse de diminuer les aides financières et les dispositifs incitatifs ? Éradiquer les « passoires thermiques » suppose de traiter tous les postes de déperdition, dont les menuiseries et tout particulièrement les fenêtres et portes d'entrée donnant sur l'extérieur. Le rapport du Centre scientifique et technique du bâtiment démontre, en effet, clairement que les travaux de remplacement d'un simple vitrage par des fenêtres performantes ont bien un impact significatif sur les consommations énergétiques finales, permettant ainsi de réaliser des économies pour le particulier. La parole

de loi de finances pour 2018 ont permis d'accompagner les contribuables et les entreprises vers la sortie de ces équipements du champ d'application du CITE. En outre, le taux réduit de 5,5 % de TVA est maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur des parois vitrées, des volets isolants, des portes d'entrée, nonobstant leur exclusion du bénéfice du CITE.

sont satisfaites dans le cadre des dispositions transitoires, puisque les contribuables qui peuvent justifier avoir engagé la réalisation de travaux d'isolation thermique de parois vitrées par l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1 juillet 2018 bénéficient des dispositions fiscales antérieures

est ainsi libellé : La parole est à Mme Colette Mélot. Les mouvements sociaux que nous connaissons ont des causes multiples. L'une d'elles est la précarité énergétique qui frappe un grand nombre de nos concitoyens les plus modestes, en particulier dans les territoires ruraux. Il n'est pas normal que les Français aient, encore aujourd'hui, du mal à se chauffer. Les amendements n II-788 et II-804 que le groupe Les Indépendants présente visent à remédier à cette précarité énergétique, tout en favorisant la transition écologique. Nous souhaitons encourager la transition des chaudières au fioul, qui coûtent cher et qui polluent, vers des chaudières plus performantes pour tous. En France, plus de 3 millions de ménages ruraux ont recours au fioul domestique comme énergie de chauffage. La part du fioul est surreprésentée parmi les ménages en situation de précarité énergétique et la hausse des prix de cette énergie devient difficilement supportable pour eux. Certes, des aides existent, comme le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE, mais elles demeurent complexes à utiliser. En pratique, seuls les ménages les plus aisés y ont recours. Nous vous présentons donc deux amendements, qui ont pour objectif de rendre ces dispositifs plus accessibles aux ménages modestes, en particulier pour ceux qui habitent dans les territoires ruraux. Quel

Sans augmenter le taux du CITE, il permet aux ménages en situation de précarité énergétique de passer à une énergie décarbonée ou de changer une chaudière à gaz de plus de quinze ans pour une chaudière de très haute performance énergétique. Il revient seulement à traduire une pratique usuelle de la part des particuliers. On nous dira que cela revient à subventionner deux fois, mais cela est nécessaire pour les ménages les plus modestes, sinon ils ne changeront jamais de chaudière. Je crois que la situation que nous traversons commande de prendre des mesures fortes en faveur de la transition énergétique des personnes les plus modestes. Il faut leur permettre de cumuler les aides publiques, l'État doit être à leurs côtés !

très justement noté que les classes moyennes étaient les grandes oubliées : elles ne pourront bénéficier ni de la surprime à la conversion des voitures ni de l'aide bonifiée pour le remplacement d'une chaudière

taux bonifié. Ainsi, lorsque la mise en oeuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1 janvier 1948, à l'obtention du label « bâtiment basse consommation basse consommation énergétique rénovation 2009 » ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l'obtention d'un label équivalent, nous proposons que le crédit d'impôt soit égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils. Quel est l'avis de la

Pour faire face en responsabilité au défi du réchauffement climatique, il nous faut décarboner notre énergie et donc développer les énergies renouvelables, parmi lesquelles l'énergie hydroélectrique.

pilotable et de faible coût. Afin d'inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, les auteurs de cet amendement proposent de faire bénéficier les nouveaux projets d'installation- je dis bien les nouveaux projets -et les projets permettant d'augmenter la capacité des installations existantes d'une exonération de taxe foncière pendant dix ans. En diminuant les charges lors des premières années d'exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets, et donc les décisions d'investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette à l'installation.

n'est pas chiffrable puisqu'elle concerne des installations qui n'existent pas encore. Elle constituerait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d'accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques. L'amendement

en pompant l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l'électricité sur le réseau en turbinant l'eau du bassin supérieur lorsque la demande électrique augmente. L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP, par nature puissantes, alors même qu'elles n'ont pas vocation à produire de l'énergie, mais à constituer une assurance pour le système électrique. Quel

des régions s'est considérablement renforcé en matière de mobilité et d'environnement. Ces dernières sont compétentes sur l'ensemble de la chaîne des transports non urbains et des transports scolaires, ainsi que sur l'intermodalité avec les agglomérations.

n'aurait en réalité aucune incidence environnementale. Par ailleurs, les régions peuvent déjà prévoir des tarifs réduits ou des exonérations en faveur des véhicules utilisant des énergies alternatives comme l'électricité, le biocarburant E85 ou le gaz de pétrole liquéfié, le GPL. Enfin, sur le plan technique, le service informatique d'immatriculation des véhicules n'est pas en mesure de gérer à court terme une progressivité de la taxe.

la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l'électricité, d'exonérer de taxe l'électricité produite par les petits producteurs, autant pour la partie autoconsommée de l'électricité qu'ils produisent que pour l'excédent revendu et réinjecté dans le réseau.

afin de permettre aux consommateurs de gaz naturel concernés par la conversion du gaz B en gaz H dans les Hauts-de-France et dont les appareils ne sont ni réglables ni adaptables de procéder à leur changement. Ce chèque serait financé par le biais du tarif d'utilisation du réseau de distribution de gaz naturel. Dans la majorité des cas, les équipements fonctionnant au gaz B peuvent être adaptés ou réglés pour pouvoir fonctionner au gaz H. Ces opérations sont prises en charge par les gestionnaires de réseau de distribution du gaz naturel et financées par les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz. dans certains cas, les équipements ne peuvent être ni réglés ni adaptés. Nous souhaitons donc mettre en place une aide spécifique sous la forme d'un chèque conversion, financé par les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz. Lors de l'examen des crédits de la mission « Écologie », dimanche dernier, dans

l'aide à la rénovation énergétique des logements. Par contre, ils pourraient jouer un rôle de conseil et orienter vers des acteurs plus à même d'aider les consommateurs sur ces sujets de rénovation thermique et énergétique. Quel est l'avis de

À défaut de garantir l'atteinte d'un haut niveau de performance énergétique globale, cette approche constitue un vrai progrès par rapport à l'approche « par élément » dont les associations rappellent le caractère inefficace. Un bouquet de travaux est ainsi un ensemble de travaux cohérents, dont la réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l'efficacité énergétique du bâtiment ou du logement. L'évolution proposée pour l'éco-PTZ dans le projet de loi de finances pour 2019 nous semble donc particulièrement inopportune en revenant sur cette conception de l'utilisation de l'éco-PTZ. Le réseau CLER, qui fédère les territoires à énergie positive, est à l'origine de cette proposition

la fiscalité de l'écologie. En attendant, je ne sais pas comment le contribuable, le citoyen, va se retrouver dans la masse de mesures hétéroclites que nous sommes en train d'adopter.

De plus, à l'issue du différé, les impositions versées par le titulaire du permis contesté sont assimilées à un paiement tardif, sanctionné d'une pénalité de 10 %. Cet amendement vise à supprimer l'obligation de constituer la garantie pour bénéficier dudit différé de paiement.

les délais de traitement des recours par le juge pouvant être longs. Il s'agit donc d'une condition habituelle en matière de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. En cas de contestation du permis de construire l'obligation pesant sur le bénéficiaire de déposer des garanties nous permet de sécuriser l'action en recouvrement à venir du comptable et ainsi de protéger les intérêts du Trésor public. La mise en oeuvre de ces garanties, si elle reste exceptionnelle, permet donc d'assurer un recouvrement effectif optimal

scolarité élevés, ou une université qui se situe loin de leur foyer, et sont contraints de souscrire un prêt étudiant, les revenus de leurs parents n'étant pas suffisants pour assurer une bonne continuité de leur scolarité. Ce prêt leur permettra de financer le prix, parfois trop élevé, de leur scolarité, leur logement, mais également les ressources scolaires exigées par les enseignants, ainsi que leurs dépenses de la vie quotidienne.

Sans remettre en cause le recours à ce type d'emprunt, cet amendement vise à supprimer le versement des intérêts pour l'ensemble des prêts étudiants, quel qu'en soit le montant, en proposant un crédit d'impôt sur ces mêmes intérêts. Cette mesure permettrait aux étudiants et aux jeunes actifs de vivre plus paisiblement cette étape de leur vie et aux familles de ne pas devoir anticiper le remboursement du prêt. L'auteur de cet amendement, qui n'a pu avoir accès au coût réel

question et à mieux prendre en compte la situation financière des jeunes actifs et de leur famille. Par ailleurs, il regrette que 200 millions d'euros de crédits de réserve de la mission

Le recentrage progressif du dispositif sur le neuf et les zones dites tendues cumulé au recentrage du « Pinel » sur ces mêmes zones et à la suppression de l'APL accession ont porté un coup majeur à la construction et la réservation de logements en France, en particulier dans les zones B2 et C. Par ailleurs, Par ailleurs, rien ne justifie de privilégier les habitants de certains territoires par rapport à d'autres. C'est un mauvais signal pour les territoires ruraux, qui ont besoin d'être attractifs. Outre qu'ils sont confrontés au vieillissement de la population, il leur sera plus difficile d'attirer de jeunes ménages et, de fait, de conserver les classes d'écoles, les bureaux de poste ou encore les cabinets médicaux. zéro dans les zones rurales doit être stabilisé sur la durée afin de maintenir le climat de confiance favorable au déclenchement des opérations d'accession. En 2016, plus de la moitié des prêts à taux zéro dans le neuf ont été distribués en zone rurale. Six opérations sur dix financées par un prêt à taux zéro ont été réalisées dans les zones B2 et C, là où les prix de l'immobilier restent encore accessibles aux ménages. Cet amendement vise à rétablir ce dispositif pour les familles modestes, qu'il s'agisse du neuf ou de l'ancien et quelle que soit la zone concernée. est également proposé de le maintenir pour des acquisitions dans l'ancien avec travaux ou lorsque l'acquéreur achète son logement social dans le cadre de la vente du patrimoine HLM voulue par le Gouvernement. Les trois présenter l'amendement n° II-85 rectifié. La diminution de moitié de la quotité du prêt à taux zéro, puis sa disparition annoncée au 31 décembre 2019 pour les opérations situées dans les communes classées B2 et C- soit 93 % des communes métropolitaines -constituent un signal alarmant pour une très grande partie du territoire français et ses habitants. Dès à présent, le nombre de prêts à taux zéro émis sur ces territoires est en diminution, impactant non seulement l'activité de construction, mais réduisant aussi les perspectives de promotion sociale des ménages à revenus modestes.

sur un zonage qu'on nous avait promis de revisiter à l'automne dernier et dont nous connaissons tous les limites. La restriction opérée l'année dernière a des effets, comme l'a dit Philippe Dallier, extrêmement négatifs sur le secteur du bâtiment et encore plus pour les

qu'il y a une vraie urgence, à la fois pour les territoires ruraux et pour le secteur du bâtiment.

Comment s'étonner, ensuite, que les gens aient un sentiment d'injustice et d'abandon ? Je vous le dis tout net, cher Marc Laménie, les amendements identiques ne vont pas dans le sens de l'équité. Ils prolongent le dispositif pour les zones B2 et C. Ils maintiennent

Même si cette mesure d'amélioration de la trésorerie des ménages apparaît être une avancée essentielle, cette initiative reste insuffisante pour soutenir pleinement la consommation des ménages ayant recours aux services à la personne et pour atteindre l'objectif d'une contemporanéité contemporanéité du crédit d'impôt relatif aux dépenses liées aux services à la personne. Seule la mise en place d'une contemporanéité effective du crédit d'impôt dès le paiement afférent à la réalisation du service est susceptible de créer l'effet de levier suffisant pour faciliter l'accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français- dont les foyers les plus modestes -, mais aussi pour accentuer la lutte contre le travail non déclaré, et dès lors l'effet attendu sur le marché de l'emploi déclaré. En effet, le premier frein à la croissance du secteur des services à la personne repose sur l'existence d'une économie illégale massive favorisée par la difficulté pour les ménages de mobiliser pendant plusieurs mois la somme d'un crédit d'impôt dont le versement est différé. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir la mise en place d'un crédit d'impôt contemporain à compter du 1 janvier 2020, à destination de l'ensemble des ménages ayant recours aux services à la personne,

Au total, le coût de cette mise en place est estimé entre 103 millions et 137 millions d'euros pour l'ensemble des TPE et entre 101 millions et 152 millions d'euros pour les PME. du titre emploi service entreprise a certes l'avantage d'être gratuit, mais il présente aussi des inconvénients. Le premier est la connaissance minimale que doit avoir le dirigeant de l'entreprise pour réaliser ses fiches de paie. Il doit en effet renseigner les horaires contractuels des salariés, les heures supplémentaires, les primes, la convention collective ... En conséquence, seuls les chefs d'entreprise déjà bien informés sont capables de recourir à ce système. De même, si le dispositif a l'avantage de la simplicité, il oblige l'entreprise à entrer dans le mécanisme du TESE. Une entreprise qui utilise déjà un autre système ne procèdera pas ainsi. L'employeur devenant collecteur d'impôt pour le compte de l'État, il est logique de lui proposer une prise en charge. Le présent amendement prévoit donc une compensation sous la forme d'un crédit d'impôt.

santé. Depuis le 1 janvier 2016, grâce à la loi ANI, une couverture complémentaire santé collective et obligatoire doit être proposée par les employeurs aux salariés de droit privé, avec l'obligation pour l'employeur de prendre à sa charge au moins 50 % de la cotisation santé. les indépendants bénéficient du dispositif dit Madelin. Cette obligation de participation des employeurs au financement de la complémentaire santé n'existe pas pas dans la fonction publique. Si certains employeurs publics font volontairement le choix de soutenir financièrement leurs agents, cette prise en charge reste volontaire et minoritaire. Ainsi, sur près de 5 milliards d'euros d'aide publique affectés à l'acquisition d'une couverture complémentaire santé, chaque année, seulement 1 % de cette somme, soit 50 millions d'euros, bénéficie aux 5,6 millions d'agents des trois versants de la fonction publique. Dans la mesure où près de 50 % des agents de la fonction publique et 75 % des agents de la fonction publique territoriale et perçoivent des revenus faibles, cette situation altère considérablement l'accès aux soins des agents de la fonction publique. Le prix élevé de la complémentaire santé est évidemment un motif de renoncement aux soins. De leur côté, les retraités ne sont pas éligibles à la majeure partie des dispositifs actuels d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé. Pourtant, les frais afférents représentent un poste de dépenses important pour les seniors, dépenses qui ont vocation à augmenter avec l'avancée en âge. Outre son caractère injuste, ce système d'aide est également complexe et peu lisible. Selon le rapport de l'IGAS du mois d'avril 2016 sur les aides fiscales et sociales à l'acquisition d'une complémentaire santé, douze dispositifs distincts existent, pour un montant total de 8,1 milliards d'euros. Ces aides sont notamment des déductions d'impôt sur les sociétés pour les entreprises, pour un montant total de 2,5 milliards d'euros, des déductions d'impôt sur le revenu pour les salariés, pour une somme de 1,2 milliard d'euros, ou encore des exemptions d'assiette de cotisations sociales patronales et salariales dans le secteur privé, pour un total de 4,3 milliards d'euros. Afin de remédier à cette situation de déséquilibre et d'harmoniser les aides octroyées, nous proposons la création d'une réduction d'impôt au bénéfice des agents et des retraités de la fonction publique pour les dépenses qu'ils engagent au titre de l'acquisition d'une complémentaire santé. Les bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS, deux dispositifs pour lesquels une réforme est en cours, ne sont pas éligibles à cette aide, car ils bénéficient déjà de dispositifs spécifiques. Les deux

privé, il est proposé la mise en place d'un crédit d'impôt pour les cotisations mutualistes acquittées par les fonctionnaires et agents publics concernés, dont les modalités seraient fixées par décret, mais dont on peut attendre qu'il vise la totalité des dépenses justifiées comme base de calcul et l'application d'un taux de 50

à une rémunération et soumise par conséquent à fiscalisation. Cela fait partie des sujets à étudier. Le rapport a été commandé à la fin du printemps dernier. Il est en cours de rédaction et devrait être rendu au Gouvernement dans les semaines qui viennent. J'ai pris l'engagement, lors de la dernière réunion multilatérale avec les organisations syndicales, que ce rapport serait immédiatement partagé avec les interlocuteurs du Gouvernement en matière de dialogue social dans la fonction publique : les représentants du collège des employeurs des

non par hostilité au principe, mais pour deux raisons : d'une part, le crédit d'impôt ne paraît pas nécessairement la bonne solution ; d'autre part, en accord avec les organisations syndicales représentatives et les employeurs publics, nous aurons le débat sur les modalités de mise en oeuvre d'une participation des employeurs au cours de l'année 2019.

disposition encourageante pour l'émigration. Ensuite, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie française, puisque le dispositif Pinel encourage les investissements immobiliers. Enfin, c'est aussi pour les Français qui sont hors de France une façon d'assurer, en partie au moins, leur retraite. Il est donc proposé que les citoyens s'établissant à l'étranger puissent garder le bénéfice du dispositif Pinel.

pour encourager le logement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, sur les zones tendues A , A et B1. La fermeture du dispositif en zones B2 et C prive les communes de ces zones, éligibles au Pinel jusqu'au 31 décembre 2017, d'un outil permettant de réhabiliter, rénover ou transformer des logements dans les centres-villes et centres-bourgs, alors même que le Gouvernement engage par ailleurs des crédits importants pour les redynamiser, dans le cadre du plan « Action coeur de ville ». Pour accompagner les élus des collectivités identifiées au sein du programme « Action coeur de ville comprises en zone B2 et C, et les doter d'un outil supplémentaire au service d'une stratégie de rénovation de leur coeur de ville, il est proposé de leur ouvrir l'accès au dispositif Pinel uniquement pour les opérations de rénovation, réhabilitation ou transformation de logements, à l'exclusion des constructions neuves. En pratique, ces opérations sont aujourd'hui peu nombreuses, car plus complexes et plus coûteuses que la construction. Le coût prévisionnel, sans être précisément quantifiable, est donc modique. À l'échelle du dispositif Pinel, la mesure proposée est marginale, mais, à l'échelle des territoires concernés, elle peut apporter une réponse déterminante à la requalification de centres-villes.

visant à appliquer, dès 2019 et non à compter de 2021, un taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de prestation de collecté séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets, afin de réduire plus rapidement encore pour les collectivités territoriales le coût de ces opérations. Quel

Cet amendement vise donc à prévoir, de manière transparente, un taux global de 10 % pour la pratique de l'équitation en centres équestres. Je rappelle que cette pratique a pu être démocratisée en France ces dernières années

par la fiscalité. À ce jour, la Fédération française d'équitation compte près de 650 000 licenciés. Il s'agit donc d'une discipline populaire, bien répartie sur l'ensemble du territoire, qu'il convient de soutenir. Enfin, pour insister sur le caractère réaliste et équitable de cette mesure, j'ajoute que l'Irlande